et de la proposition de loi organique, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (proposition n°

Nous parlons de droit électoral, l'une des matières les plus sensibles politiquement que nous ayons à traiter. Il aurait été facile de raisonner par postures et de refuser de construire ensemble : cela n'a pas été le cas. Il est vrai que ces textes répondent à des impératifs. C'est en se saisissant des remarques réalisées par le Conseil constitutionnel après les élections législatives qu'Alain Richard a conçu ces propositions de loi, qui permettent de corriger quelques zones d'ombre de notre droit électoral et d'aller vers plus de clarté et d'homogénéité. Ainsi, ces textes sont animés par la volonté de rendre notre droit électoral plus équitable et de combler les manquements et les failles que nous constatons à l'occasion des scrutins. La première avancée réside dans l'homogénéisation des règles de campagne électorale. Aujourd'hui, une divergence entre les parties législative et réglementaire du code électoral provoque une incohérence dans ces règles. Ainsi, si les tractages, collages ou publications sur les réseaux sociaux sont logiquement interdits à partir de la nuit entre le vendredi et le samedi du jour qui précède le vote, il n'en est pas de même pour les réunions publiques qui sont théoriquement autorisées le samedi qui précède le jour du scrutin. Il y avait là quelque chose d'anormal et la proposition de loi permet de résoudre ce paradoxe. Ainsi, le code électoral sera désormais homogène et toutes les opérations électorales, sans exception, seront interdites à partir de la veille du scrutin à minuit, c'est-à-dire dans la nuit du vendredi à samedi précédent le dimanche de scrutin. Désormais, les candidats seront sur un pied d'égalité et ne pourront plus faire valoir cette ambiguïté du droit. La deuxième grande avancée concerne les bulletins de vote. Avec les nouveaux usages, les candidats aux élections ont montré que leur imagination en termes de de design des bulletins ne connaissait pas de limite. Ce fait a été notamment observé avec l'apparition de plus en plus fréquente de photos. Si cet usage en soi ne pose pas de difficultés, il était curieux qu'il soit interdit de faire figurer sur les bulletins de vote le nom de quelqu'un qui n'est pas candidat, mais qu'il soit possible de faire apparaître la photo d'un non-candidat. Grâce aux nouvelles dispositions prévues, il sera désormais impossible de faire figurer sur les bulletins des photos de tiers : seuls les candidats pourront être représentés. De même, si le principe d'interdiction de faire figurer le nom de quelqu'un qui n'était pas candidat sur un bulletin de vote existe, il était l'objet d'une interprétation assez souple, voire divergente. Cela pouvait prêter à confusion et conduire à des abus. Aussi est désormais explicitement affirmée l'interdiction de faire paraître le nom d'un tiers sur un bulletin. Je crois qu'il s'agit de principes sains et utiles. Nous ne devons pas courir le risque d'induire les électeurs en erreur : désormais, les bulletins viseront les seuls candidats, rien que les candidats. Ensuite, les textes que nous examinons vont au-delà des recommandations du Conseil constitutionnel et permettent des avancées supplémentaires. Je pense en particulier aux obligations et aux délais de déclaration pour demander un remboursement des frais de campagne. Tout cela demeurait un peu flou, et les recommandations de la Haute Autorité pour la

soulèvent des questions pertinentes dont nous comprenons la logique, il est essentiel que la navette parlementaire puisse s'achever avant les élections municipales, afin que les dispositions prévues puissent s'appliquer le plus rapidement possible, notamment au prochain scrutin. D'autres travaux pourront être menés ensuite. Notre droit électoral peut encore évoluer, encore s'améliorer. Nous y sommes ouverts et je veux saluer le travail mené par Alain Richard, M. le rapporteur et les parlementaires sur ces sujets. Il me semble néanmoins important que les dispositions de ces propositions de loi soient assurément prêtes à être appliquées pour les prochaines élections municipales. La parole

chers collègues, nous débattons en seconde lecture des deux propositions de loi ordinaire et organique déposées par Alain Richard, qui clarifient diverses dispositions du code électoral. J'en rappelle les deux objectifs : clarifier les règles de financement des campagnes électorales, d'une part, mieux encadrer la propagande et les opérations électorales, d'autre part. L'Assemblée nationale a adopté ces propositions de loi le 24 septembre dernier. S'efforçant de respecter l'équilibre trouvé par le Sénat, elle a voté conformes six articles de la proposition de loi et un article

Afin d'adapter notre droit électoral aux nouvelles pratiques politiques, la proposition de loi permet aux candidats et aux partis politiques d'utiliser des plateformes en ligne pour recueillir les dons des personnes physiques, la traçabilité des transactions financières étant renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Concernant la définition des menues dépenses que le candidat peut régler directement sans passer par son mandataire financier, nos collègues Roger Karoutchi et Françoise Laborde avaient souhaité fixer dans la loi le montant maximal de ces dépenses 10 % du montant total du compte de campagne et à 3 % du plafond des dépenses électorales. Je les remercie très sincèrement de cette initiative, qui permet d'ouvrir un débat important pour l'ensemble des candidats et de clarifier l'intention du législateur.

menues dépenses. Elle a étendu l'obligation d'établir un compte de campagne à l'ensemble des candidats aux élections européennes, même lorsqu'ils ont réuni moins de 1 % des suffrages exprimés. En effet, avec le rétablissement d'une circonscription unique, une liste de candidats aurait pu mener campagne campagne à l'échelon national et recueillir jusqu'à 226 000 voix sans déposer de comptes de campagne, ce qui paraît incompatible avec la nécessaire transparence du scrutin. Les députés n'ont pas adopté de modification majeure quant au déroulement de la campagne électorale ou à la propagande. Ils ont notamment conservé l'interdiction, pour plus de sécurité juridique, d'organiser des réunions électorales la veille du scrutin. Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a souhaité préciser le calendrier des campagnes électorales, principalement pour les élections législatives, en en réduisant le délai de vingt à quatorze de vingt à quatorze jours. Les députés ont également conservé la possibilité pour le maire ou, à défaut, le préfet de procéder à la dépose d'office des affiches apposées hors des emplacements réservés. Ce point nous a

l'Assemblée nationale a adopté une position de compromis en autorisant la mention du nom d'un tiers pour les seules villes à secteurs et arrondissements- Paris, Lyon, Marseille -, ainsi que la photographie des candidats. Une telle perspective avait été évoquée dans cet hémicycle. S'agissant des inéligibilités, les propositions de loi permettent de clarifier le droit en vigueur en rappelant qu'une simple erreur matérielle d'un candidat ne doit pas empêcher ce dernier de se présenter aux scrutins suivants. Nous donnons ainsi plus de sécurité juridique aux candidats, ce qui me semble essentiel. Avec l'accord du Gouvernement, nous avons également adapté le régime d'inéligibilité des préfets et des sous-préfets, notamment pour éviter qu'ils ne puissent se présenter aux élections municipales dans les jours qui suivent leur admission à la retraite.

L'inéligibilité s'appliquant à compter de la décision définitive du juge de l'élection, l'effet de la sanction varie d'un candidat à un autre, en fonction de la durée d'instruction de son dossier. En première lecture, le Sénat avait proposé d'autoriser le juge de l'élection à moduler la durée d'inéligibilité. L'objectif était de s'intéresser au « point d'arrivée » de l'inéligibilité pour que des candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes scrutins. L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette ingénieuse proposition, laissant donc perdurer le droit en vigueur. Il est vrai que, malgré son ingéniosité, cette mesure soulevait quelques difficultés en matière d'égalité entre les personnes concernées Je remercie chaleureusement Alain Richard d'avoir déposé un amendement non seulement pour poursuivre la réflexion sur ce sujet, mais surtout pour nous permettre de préciser l'intention du législateur à l'égard du juge des élections. Afin que ces deux propositions de loi de clarification nécessaire du droit électoral puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais, la commission des lois les a adoptées sans modification.

Sans revoir l'ensemble de ce code, les deux textes de notre collègue Alain Richard ont des objectifs sains. Ils s'inspirent directement des observations formulées par le Conseil constitutionnel sur les dernières élections législatives. Toutefois, ils concernent l'ensemble des élections, y compris les élections locales. Je me réjouis tout particulièrement des efforts de clarification de ces textes, à la fois techniques et pragmatiques. Ces propositions de loi ont par la suite été enrichies en commission des lois et en séance au Sénat, en première lecture. Au cours de leurs travaux, nos collègues députés se sont efforcés de respecter l'équilibre des propositions de loi adoptées par le Sénat et de les enrichir. Ils ont ainsi étendu l'obligation d'établir un compte de campagne à l'ensemble des candidats

En première lecture, le Sénat a autorisé le juge de l'élection à moduler la durée des inéligibilités, l'objectif étant que des candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes scrutins. L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette proposition. Le droit en vigueur sera donc maintenu, faute de consensus. Toutefois, ces deux textes constituent un bon compromis entre nos deux assemblées.

les propositions de loi, ordinaire et organique, qui nous sont soumises aujourd'hui en deuxième lecture. Ces textes corrigent, à la suite des observations formulées par le Conseil constitutionnel au lendemain des élections législatives de 2017, de nombreuses imperfections qui émaillent notre droit électoral, en particulier à l'échelon local. Ils clarifient opportunément le le contrôle des dépenses électorales et des règles d'inéligibilité. Enfin, ils améliorent l'encadrement de la propagande électorale et des opérations de vote. On ne peut que s'en féliciter, tant la fiabilité des processus électoraux conditionne la bonne santé de la vie démocratique. Plus généralement, ces deux propositions de loi participent de l'adaptation de notre législation aux défis de la modernité. J'en veux pour preuve l'article 1 A, qui devrait permettre demain la perception de dons en ligne, subordonnés à des conditions, notamment de traçabilité, de nature à garantir garantir aux électeurs l'intégrité du processus électif. Nous saluons également la suppression de l'obligation, parfois onéreuse, de recourir à un expert-comptable pour les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages et dont les recettes et dépenses n'excèdent pas un certain montant. C'est là, pour les petits candidats, une simplification bienvenue de leurs démarches administratives. Nous saluons encore l'harmonisation des délais relatifs à la tenue des réunions électorales. En prohibant de manière uniforme ces réunions à compter de la veille du scrutin, le texte prémunit les candidats contre le risque de de contentieux, sécurisant ainsi le bon déroulement de leur campagne. Nous nourrissons néanmoins quelques regrets ... Nous regrettons ainsi que l'Assemblée nationale ait écarté l'article 1 A, A, qui autorisait un candidat à régler directement des dépenses inférieures à des plafonds fixés par la loi. Combien de candidats connaissent, en effet, ce problème ? Il n'eût pas été inutile de préciser dans la loi le champ de ces « menues dépenses Les difficultés rencontrées par les candidats pour contracter un emprunt auprès des banques ne sont pas davantage traitées dans ces textes. Or l'octroi de prêts bancaires aux candidats à une élection est de plus en plus étroitement encadré par la législation électorale. Le problème s'est, hélas !, de nouveau présenté lors des dernières élections européennes. Nous déplorons également le maintien pur et simple du droit ordinaire et organique en vigueur concernant le point de départ de la peine d'inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales ou pour fraude électorale. Si nous pouvons comprendre les griefs de nos homologues députés, liés en particulier à la rétroactivité de la mesure sur les mandats en cours, nous aurions aimé qu'une autre solution soit proposée. Celle-ci aurait pu consister, par exemple, à ouvrir la faculté pour le juge de moduler la peine, de façon à prendre en considération le calendrier électoral à venir. Toujours est-il que le compromis trouvé, tel qu'il résulte des travaux des deux assemblées, est globalement satisfaisant,

la célérité avec laquelle ont prospéré ces propositions de loi. Celle-ci doit nous inspirer en vue des prochains textes que nous aurons à examiner. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste est favorable à ces propositions de loi, qui, tout en modernisant utilement notre droit électoral, en suppriment de nombreuses dispositions, devenues au fil du temps sources d'incohérences et de complexité. La parole

Ces textes sont pour l'essentiel consacrés aux conditions de financement des campagnes et au contrôle des opérations électorales. Parmi les mesures de simplification intéressantes, je relèverai celles qui permettent d'utiliser des plateformes en ligne pour recueillir les dons des personnes physiques. mesure constitue une dérogation au principe selon lequel toutes les opérations financières liées à la campagne doivent transiter directement par le compte du mandataire, mais, compte tenu des évolutions de notre époque et du rôle croissant joué par le numérique dans notre société et en politique, une telle dérogation me paraît judicieuse. D'autres mesures utiles concernent l'harmonisation sur le point de départ des délais de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou encore la simplification des démarches des candidats dans le cadre de la tenue du compte de campagne. Enfin, je ne saurais omettre la codification, à l'article 6 de la proposition de loi ordinaire, de ce qui relevait jusqu'à présent de la seule tradition républicaine le principe d'immutabilité du régime électoral et du périmètre des circonscriptions dans l'année précédant toute élection. L'Assemblée nationale a donc respecté pour l'essentiel l'équilibre de ces mesures d'origine sénatoriale.

Ceux-ci ont jugé préférable de supprimer l'article 1 de la proposition de loi ordinaire, introduit à la suite de l'adoption de l'amendement de notre collègue Roger Karoutchi. Cet article portait sur le régime juridique des « menues dépenses », ces dépenses que le candidat peut régler directement, sans passer par le mandataire financier. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a jugé que l'existence de ces menues dépenses représentait une simple tolérance, qu'il ne fallait pas transformer en règle. Cependant, en écartant cette disposition,

Malgré ces deux ombres au tableau, et à l'approche des échéances électorales, le rapporteur et la commission ont choisi de recommander le vote conforme d'un texte qui comporte des avancées utiles. Je m'associe à cette position, mais non sans regrets, car la suppression de ces deux mesures par l'Assemblée nationale constitue à mes yeux un recul. C'est aussi le sentiment de plusieurs de mes collègues de la commission des lois, comme ils l'ont indiqué hier matin.

toutefois décidé de ne pas déposer d'amendements lors de cette ultime lecture, considérant d'abord qu'il était utile de rechercher

est d'éviter qu'une simple erreur matérielle sans volonté de fraude n'entraîne l'inéligibilité d'un candidat. Or la jurisprudence est constante

La proposition de loi confirme ainsi que les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ont l'interdiction d'apporter leur garantie aux prêts contractés par les candidats. C'est là une clarification nécessaire.

La proposition de loi élève au niveau législatif les règles encadrant l'ouverture et la fin des campagnes électorales, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale.

texte. Enfin, et je terminerai par ce point, il est bénéfique d'instaurer dans la loi l'interdiction de modifier les règles électorales ou le périmètre des circonscriptions l'année précédant le premier tour de scrutin.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la seconde lecture d'un texte législatif est aujourd'hui devenue une rareté, presque un objet de curiosité parlementaire. Les deux textes que nous examinons aujourd'hui entrent dans cette catégorie. Ils nous reviennent dans le cadre d'une véritable navette, c'est-à-dire à l'issue d'un dialogue constructif entre les deux assemblées. Mon groupe salue bien sûr une nouvelle fois l'initiative prise par notre collègue Alain Richard, ainsi que le travail méticuleux de M. le rapporteur, Arnaud de Belenet.

Comme nous l'avions déjà souligné, cette disposition aurait pourtant contribué à réduire les risques juridiques pour les candidats, tout en limitant les sources de contentieux et d'inéligibilité. Les autres dispositions restant en discussion nous paraissent aller dans la bonne direction, comme je l'avais déjà relevé lors de la première lecture, qu'il s'agisse de la simplification des règles comptables, des règles de propagande électorale ou des règles de délai. Le rapporteur l'a lui aussi souligné : les modifications apportées par les députés, hormis la suppression de notre amendement, sont finalement secondaires et confortent la philosophie générale du texte. L'allongement de la durée d'inéligibilité des membres du corps préfectoral en particulier emporte notre approbation, mon groupe défendant depuis longtemps le renforcement de l'équité entre candidats par l'établissement de règles d'inéligibilité plus strictes pour les personnes disposant d'un avantage Par ailleurs, l'obligation actuelle de déclaration d'inéligibilité d'un candidat « en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » devient une possibilité. Il s'agit d'une évolution pragmatique et simplificatrice qui évitera des sanctions disproportionnées. Toujours en matière de simplification des règles, nous ne pouvons que souscrire à l'allégement des obligations de dépôt de compte de campagne, ou encore à l'extension de la dérogation du recours à un expert-comptable. Afin de parvenir à une plus grande équité entre candidats, nous soutenons évidemment la mise en cohérence des règles relatives à l'organisation des réunions électorales ou à la clarification des règles de délai et de forme des déclarations de situation patrimoniale. Enfin, la codification de la règle voulant que l'on ne change pas le mode de scrutin ou le périmètre d'une circonscription durant l'année qui précède le scrutin, qui était jusque-là un usage républicain, est certainement la bienvenue,

De façon plus générale, nous considérons que de nombreuses annulations de scrutins ont pour origine la grande complexité des règles applicables et non la moralité douteuse des candidats. Notre propension au pointillisme administratif crée souvent des barrières d'entrée qui découragent les vocations des candidats potentiels les moins bien informés. Nous devons donc progresser dans l'équilibre entre simplification des règles et renforcement de notre législation relative au financement de la vie démocratique.

Il faudra véritablement se pencher un jour sur cette question, rendue problématique par la trop grande complexité des règles de domiciliation électorale.

Cela étant dit, le groupe RDSE considère que l'initiative de notre collègue Alain Richard aurait pu être l'occasion d'un toilettage plus ambitieux du code électoral, l'occasion surtout d'engager une réflexion plus approfondie sur la modernisation du financement de la vie politique, et plus largement, de notre démocratie. Pour autant, nous n'avons pas déposé d'amendements, car nous considérons qu'il est préférable que ces deux textes soient rapidement adoptés, afin de permettre leur entrée en vigueur en vue des prochaines élections municipales. Vous l'aurez compris, nous les voterons. La parole

à ces deux propositions de loi : la clarification de la date de fin de campagne, tous éléments confondus ; les améliorations concernant le contenu du bulletin,

Cet amendement serait naturellement adopté dans l'enthousiasme général des foules présentes. Mais j'ai bien entendu M. le rapporteur,

étant entendu que je considère que, dorénavant, j'ai une créance sur de futurs amendements ! L'amendement

singulier et rare pour être souligné ! Je veux simplement, non pas compléter les propos d'Alain Richard, mais mettre en exergue

une préconisation presque explicite du Conseil constitutionnel, cette solution ne peut prospérer, car elle pose d'évidents problèmes de rétroactivité : de la légalité des décisions prises entre temps ? des indemnités ? Même si

de conforter la conviction de ceux qui ne voudraient pas revenir à cette fausse bonne idée, point de départ de nos travaux sur ce sujet.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Je vous invite, mes chers collègues, à vérifier que votre carte de vote est bien insérée dans votre terminal.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la question des arrêts cardiaques nous concerne tous. Chaque année, 40 000 personnes meurent en France d'un arrêt cardiaque inopiné

Ces chiffres démontrent deux choses : une urgence à agir et une urgence à former. C'est l'objet même de la proposition de loi déposée par Jean-Charles Colas-Roy à l'Assemblée nationale. Ce texte n'appelle pas aux débats partisans, mais à la responsabilité de toutes et tous. C'est d'ailleurs cet esprit qui avait prévalu à l'Assemblée nationale, où le texte avait été adopté à l'unanimité. J'aimerais revenir sur les fondements et les objectifs de ce texte. Dès son élection, le Président de la République avait fixé un objectif aussi nécessaire qu'ambitieux : former 80 % de la population aux gestes qui sauvent d'ici à dix ans. C'est d'autant plus essentiel que 70 % des attaques cardiaques se déroulent devant des témoins et que chaque minute compte. veux vous en donner une idée précise : sans massage cardiaque, les chances de survie s'amenuisent de 10 % par minute. Au-delà de trois minutes sans massage, les lésions provoquées sont généralement irréversibles. Au-delà de dix minutes, les chances de survie sont pratiquement nulles.

Aussi, augmenter le nombre de personnes formées et capables d'intervenir vite en cas de détresse permettra de sauver des vies. À nouveau, des chiffres seront plus parlants : si nous atteignons l'objectif fixé par le Président de la République, nous augmenterons le taux de survie de 3 % à 10 % et sauverons 3 000 vies chaque année. Bien sûr, ces chiffres sont théoriques, ils n'en demeurent pas moins parlants. Cette proposition de loi nous permet d'aller dans le bon sens. Dans le texte issu des travaux de la commission

Il s'agit d'une mesure importante, car aujourd'hui une personne qui pratique un massage cardiaque sur une victime n'est pas protégée par le droit et peut être exposée à des poursuites. Le sauveteur occasionnel, c'est-à-dire la personne qui pratique un geste de premiers secours, doit bénéficier d'une protection et de reconnaissance pour son geste. Par ailleurs, nous devons responsabiliser les Français par tout moyen ; c'est pourquoi l'article 11 de la proposition de loi renforce les peines en cas de vol ou de détérioration d'un défibrillateur. Le Sénat a beaucoup transformé le texte issu de l'Assemblée nationale. Si je comprends parfaitement sa volonté de législateur d'opérer une séparation rigoureuse des mesures législatives et réglementaires, je crains qu'il ne soit allé un peu trop loin, en supprimant quelques-uns des effets utiles du texte. Je ne prendrai qu'un exemple : son changement de titre. Avoir remplacé les « gestes qui sauvent » par « les premiers secours » implique un changement et une réduction assez importante du champ d'application du texte.

Il me paraissait donc utile de maintenir leur mention dans le nom de la proposition de loi afin de continuer à y faire référence. Il importe par ailleurs que la notion de collaborateur occasionnel du service public, consacrée par la jurisprudence administrative, puisse trouver à s'appliquer non seulement au au sauveteur occasionnel, mais aussi à d'autres acteurs du secours. En ce sens, j'émettrai un avis favorable sur l'amendement déposé par le groupe La République En Marche, qui vient consolider la rédaction de l'article 1 de cette proposition

pour notre prévention et contre les risques d'accident cardiaque. Encore une fois, nous aurons l'occasion de débattre de cette articulation entre le statut de sauveteur occasionnel et celui, jurisprudentiel, de collaborateur

l'arrêt cardiaque subit demeure une des causes de mortalité les plus importantes et méconnues du grand public. En France, entre 40 000 et 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque chaque année, soit quinze fois plus que le nombre de morts sur les routes. pire est de ne rien faire, comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, puisque le délai d'intervention a un impact très significatif sur les chances de survie de la victime. Sans prise en charge immédiate, plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals. fois sur dix, ces arrêts surviennent devant témoins, mais seulement 40 % de ceux-ci font les gestes de premiers secours. La conséquence triste, mais logique, est qu'en France le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas les 8 %, ce taux étant quatre à cinq fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent. Face à ce constat, plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises. Je fais ici référence à la loi du 13 août 2004 rendant obligatoire l'apprentissage des gestes qui sauvent à l'école. Je fais également référence à la loi du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, qui est issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Leleux. Je fais enfin référence à la loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque, issue quant à elle d'une proposition de notre collègue Jean-Pierre Decool. C'est dans cette perspective que se situe la proposition de loi déposée par notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Son objectif est à la fois clair et louable porter l'attention sur ce sujet majeur et favoriser les interventions, d'une part, en formant la population aux gestes qui sauvent et, d'autre part, en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention. Partageant pleinement ces objectifs, la commission des lois a examiné le texte de l'Assemblée nationale au travers d'un crible rigoureux afin d'en garantir l'efficacité. Elle n'a donc pas hésité à écarter des dispositions qui ne relèvent pas du domaine que la Constitution confie à la loi, qu'elles fussent soit de nature réglementaire, soit dépourvues de portée normative. Je me félicite d'ores et déjà que la méthode proposée ait reçu l'assentiment de notre assemblée, puisque les amendements déposés ne portent que sur des points techniques précis et ne tendent pas à ce que le texte ne tendent pas à ce que le texte retrouve son champ initial. La commission des lois a tout particulièrement porté son attention sur l'article 1 de la proposition de loi qui tend à créer un statut de « citoyen sauveteur » afin de mieux protéger les personnes venant en aide de manière volontaire et bénévole aux victimes d'une urgence vitale. Nous avons souhaité réécrire cette disposition afin de redéfinir les conditions d'intervention des sauveteurs dans des termes plus juridiques. Ainsi, la commission des lois a remplacé l'expression de « citoyen sauveteur » par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole » qui est plus appropriée au concours apporté à l'exercice d'un service public. La commission des lois a souhaité conserver du texte transmis la référence au régime jurisprudentiel de collaborateur occasionnel du service public, les atténuations de responsabilité pénale et le régime spécial de responsabilité civile applicable aux sauveteurs. Toutefois, elle a souhaité apporter une correction de nature à l'exonérer pour tous les préjudices qu'il pourrait causer lors de son intervention, sauf faute lourde ou intentionnelle, et pas seulement pour ceux causés à la personne secourue elle-même. De plus, j'ai souhaité tenir compte d'une partie des remarques soulevées par l'amendement déposé par le groupe La République En Marche. En ce sens, l'amendement que je vais vous présenter réintroduit les obligations d'appeler les secours et de prendre les premières dispositions pour toute personne, personne, et non pas pour les seuls sauveteurs occasionnels. En revanche, il ne semble pas opportun d'élargir le champ de la proposition de loi à tous les acteurs de la sécurité civile, comme le prévoit l'amendement du groupe La République En Marche, puisque l'objectif est bien de consacrer un régime spécial pour les sauveteurs occasionnels et eux seuls. Par ailleurs, la commission des lois a approuvé les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi qui tendent à consolider la liste des personnes autorisées à accomplir les actes de sensibilisation au secourisme. Elle a seulement souhaité y inclure certains services des établissements de santé. En effet, beaucoup d'entre eux détiennent les compétences nécessaires pour assurer une formation au secourisme. Enfin, la commission des lois s'est également montrée favorable aux dispositions de l'article 11 tendant à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs. Les modifications qu'elle a apportées ont pour seul objet d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale. Vous le voyez, mes chers collègues, la commission des lois a souhaité ne garder dans ce texte que des dispositions efficaces et effectives. Par l'amendement que je vais vous présenter, elle a également souhaité faire un pas

Si des dispositions bien faites sont indispensables, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour lutter contre les arrêts cardiaques. Je pense sincèrement que la nécessité de se former aux premiers secours découle d'une obligation morale et civique pour toute personne, notamment celles qui ont la charge d'en encadrer d'autres, dans quelque contexte que ce soit. Il devrait s'agir là d'un réflexe que nous devrions tous avoir. La parole

nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à créer le statut de citoyen sauveteur, à lutter contre l'arrêt cardiaque et à sensibiliser aux gestes qui sauvent. Cette

des pompiers, souvent volontaires, des policiers, des urgentistes, prennent des risques pour veiller sur leur prochain et porter secours à celui ou celle qui se trouve en danger. Nous ne devons pas banaliser l'engagement quotidien de ces héros. Leur courage fait entrer l'exceptionnel dans l'ordinaire. Au contraire, nous devons plutôt nous interroger, nous autres citoyens qui ne prenons pas de tels risques au quotidien. Nous devons nous interroger pour savoir si, à notre échelle, nous serions en mesure de suppléer ces héros, dans le cas où nous serions seuls à pouvoir intervenir. C'est tout l'intérêt que revêt, à mes yeux, cette proposition de loi. Elle vise à faciliter et à sécuriser la capacité de tout un chacun à faire le bon geste au bon moment. Évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu, mais qui pense que nous ne devrions pas, collectivement, relever encore un peu notre niveau d'exigence pour prévenir au mieux ces risques, auxquels chacun d'entre nous est exposé L'ambition de cette proposition de loi est noble ; cela ne fait aucun doute. Absolument ! Mais je partage l'avis de la commission : la version initiale contenait d'importants risques juridiques. C'est notamment le cas pour l'article 1. La nouvelle mouture du texte permettra de mieux sécuriser les citoyens qui portent assistance, de façon occasionnelle et bénévole, à un autre citoyen, tout en garantissant leur protection juridique. Ce serait le comble que de susciter doutes et appréhensions, alors que nous souhaitons encourager la prise d'initiative Je me réjouis également que les sanctions portant sur les vols de défibrillateurs cardiaques soient renforcées. J'y vois le complément utile de la loi issue de la proposition de notre collègue Jean-Pierre Decool qui a permis de développer l'accès aux défibrillateurs automatisés externes, en rendant leur présence obligatoire dans certains lieux. Il s'agit d'équipements dont nous devrions être systématiquement entourés et les vols de tels matériels constituent, dans cette optique, une atteinte grave à la solidarité et à la cohésion nationales. Comment croire en la bienveillance collective si l'on découvre, trop tard, que l'équipement indispensable à la survie d'un citoyen a été subtilisé pour de petits profits ? L'État doit se montrer particulièrement ferme sur ce sujet. Fermeté de la puissance publique, engagement bienveillant des citoyens au service de leurs proches : l'État ne peut pas tout et chacun doit se mobiliser sans attendre des solutions qui viennent d'en haut. Je partage cette vision de la société, sans verser pour autant dans l'angélisme. Je mesure ce qu'elle implique d'exigence collective, mais je crois qu'elle nous permettra de nous élever tous ensemble. Chacun le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ne nous laissons pas abuser par des ambitions qui flattent notre courage, mais nous contraindraient de façon excessive. Se mettre au service de tous n'implique pas de devenir l'obligé de chacun. Je pense que le Sénat a sagement amendé ce texte, qui se trouve désormais réduit à ses propositions les plus essentielles. Il conserve à mes yeux sa pertinence et atteint mieux encore son objectif initial. Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur du texte, tel qu'il a été retravaillé par la commission des lois.

». C'est exact, la commission des lois l'a démontré : ce sujet est déjà traité par ailleurs. C'est la raison pour laquelle la commission a sensiblement

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, 8 %, c'est le taux de survie en France d'une personne victime d'un arrêt cardiaque inopiné. Dans un pays comme le nôtre qui se distingue par une large accessibilité aux soins et une médecine de qualité, ce chiffre ne peut que nous scandaliser, surtout quand on le compare à celui des pays anglo-saxons et scandinaves, où il est trois à quatre fois plus élevé. Dans ce contexte, nous pouvons dire que les dispositions de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sont des mesures de santé publique. Elles visent à inciter nos concitoyens à se former et surtout à ne plus hésiter à agir, lorsqu'ils sont témoins d'un tel accident. Je ne reprendrai pas les chiffres déjà cités, mais il faut savoir que, lors d'un arrêt cardiaque inopiné, pour chaque minute qui s'écoule sans pratique d'un massage cardiaque, ce sont 10 % de chances de survie en moins pour la victime. Quand on sait qu'en France les secours mettent en moyenne treize minutes pour arriver, on comprend que les premiers soins prodigués par un témoin, notamment le massage cardiaque, peuvent sauver une vie. Cette proposition de loi veut donc donner, ce qui est bienvenu, un véritable statut à ces héros du quotidien. L'article 1 permet de graver dans le marbre de la loi le statut de ces sauveteurs occasionnels et bénévoles, le terme de citoyen ayant été jugé à juste titre inapproprié par notre commission des lois. Ce statut Ce statut permettra d'inscrire dans la loi une jurisprudence existante et de protéger ainsi juridiquement « quiconque porte assistance de manière spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent Avec cette formulation, le texte issu des travaux de la commission des lois a vocation à englober toute sorte d'accidents graves, et pas seulement l'arrêt cardiaque, renforçant ainsi la protection conférée. L'atténuation de la responsabilité pénale en cas de délit non intentionnel lors de l'intervention du sauveteur bénévole et l'exonération de tous les préjudices qu'il pourrait causer, sauf bien évidemment en cas de faute lourde ou intentionnelle, sont à la fois de justes contreparties au service rendu et des incitations pour lutter contre une inaction mortifère. S'agissant des mesures de sensibilisation aux gestes qui sauvent prévues dans le texte initial, la commission des lois a supprimé une grande partie d'entre elles, car elles existent déjà ou relèvent du domaine du règlement. Je partage cette volonté de ne pas faire de l'affichage, mais de prendre des mesures concrètes. Néanmoins, si la sensibilisation et la formation des écoliers et des salariés existent déjà, elles mériteraient certainement une meilleure visibilité et même une plus grande publicité afin que tous les citoyens, quel que soit leur âge ou leur profession, soient conscients de l'importance de se former régulièrement, et surtout de l'importance d'agir.

Cette formation favorisera la prise en charge rapide d'un sportif en situation de malaise cardiaque. Enfin, le renforcement des sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation des défibrillateurs cardiaques aura, je l'espère, une vertu comminatoire et permettra d'affirmer la fermeté de l'État contre ces délits odieux qui mettent en danger la vie de nos concitoyens. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce texte ne peut que faire l'objet d'un compromis, tant le sujet qu'il traite est grave. Néanmoins, j'attire l'attention du Gouvernement sur l'importance de la sensibilisation et de la formation continue aux gestes de premiers secours. La peur de mal faire et l'incompétence favorisent l'inertie. De l'audace, toujours de l'audace », disait le révolutionnaire Georges Danton. Il faut espérer que ce texte, qui sera voté par le groupe du RDSE, en donnera un maximum à nos concitoyens ! Très bien

sa proposition de loi comporte un caractère de nécessité à au moins deux égards. Déjà, parce qu'elle met en lumière un fait essentiel : l'arrêt cardiaque inopiné n'a rien d'une fatalité et, en aucun cas, il ne doit être perçu comme tel. Loin d'être un facteur de résignation, le taux de survie extrêmement faible aux arrêts cardiaques inopinés en France, de l'ordre de 3 % à 4 %, met au jour les insuffisances de notre droit. Ce taux de survie résiduel doit, me semble-t-il, nous faire l'effet d'une injonction à agir. J'en veux pour preuve qu'un tiers des Français seulement est formé aux comportements qui sauvent. Proportion terriblement insuffisante au regard de l'objectif de 80 % fixé par le Président de la République. En instituant un régime de responsabilité protecteur pour le citoyen portant assistance à une personne en situation de péril grave et imminent, mais aussi en renforçant les dispositifs de sensibilisation aux gestes qui sauvent, cette proposition de loi présente un double intérêt elle s'attaque d'abord à un problème majeur de santé publique ; elle organise ensuite, sur un plan secondaire, mais non moins fondamental, un vecteur de solidarité entre les citoyens. Face au risque d'arrêt cardiaque inopiné, personne n'est épargné. Face au risque d'arrêt cardiaque inopiné, tout le monde peut intervenir. Chaque citoyen constitue un maillon de la chaîne de survie. Et chaque citoyen peut être appelé en toutes circonstances à se draper dans les habits du sauveteur. Et cela, bien avant l'arrivée des secours médicalisés. Favorisons donc ces démarches, que je ne me refuse pas à caractériser de providentielles, et renforçons le cadre juridique par lequel cette faculté d'assistance réciproque, au fondement de notre pacte social, pourra s'exercer Mes chers collègues, la nécessité de ce texte a été admise par un consentement unanime. D'abord, à l'Assemblée nationale ; ensuite, je crois pouvoir le dire, au Sénat. Offrons-lui donc l'assise juridique qui en garantira une bonne application Nous avons jugé la rédaction retenue par la commission plutôt satisfaisante. Elle crée notamment un régime protecteur pour les citoyens procédant bénévolement aux premiers secours sur autrui et elle renforce les peines prévues pour vol ou dégradation de défibrillateur. Il nous apparaît cependant opportun d'aller plus loin. Nous vous proposerons, lors de l'examen des amendements, d'inscrire dans le marbre de la loi la théorie du collaborateur occasionnel du service public de la sécurité civile, applicable à toute personne concourant à la sécurité civile et pas seulement à celle qui porte assistance à une personne en situation apparente de péril grave et imminent.

La commission a réécrit et précisé la définition imaginée par l'Assemblée nationale dans les termes que vous avez rappelés, madame la rapporteure,

personnels des services de l'État et militaires investis de missions de sécurité civile. Apparemment, tous les professionnels de santé semblent s'accorder sur le bien-fondé du statut qui nous est proposé,

cela n'étonnera personne ! -, l'article 11 qui renforce les peines contre les vols, destructions ou dégradations de défibrillateurs cardiaques pour les porter à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

En revanche, par courage ou par instinct, toujours avec une profonde humanité, ils portent secours et assistance à une personne qu'ils ne connaissent pas et dont ils ignorent souvent tout. Les histoires de ces citoyens qui refusent de passer leur chemin et qui voient dans les difficultés de l'autre un peu d'eux-mêmes nous touchent et nous bouleversent, car elles révèlent ce que nous avons de meilleur en nous : un refus de l'individualisme pourtant si prégnant de nos jours et une forme d'abnégation qui force le respect.

40 000 à 50 000 personnes décèdent de mort subite, que l'on appelle aussi arrêt cardiaque inopiné. Le nombre de ces décès est dix fois supérieur à celui des accidents de la route. Cela donne une idée assez précise de l'enjeu. Il nous appartient aujourd'hui de démontrer que ces décès ne sont pas une fatalité, mais que nous pouvons contribuer à mieux les combattre en permettant à chacun d'entre nous d'être des sauveteurs potentiels. Le citoyen ou le témoin présent au côté de la victime qui s'effondre est le premier maillon indispensable, et souvent vital, de la chaîne de secours, car chaque minute compte. En effet, sur ces 40 000 à 50 000 décès annuels, 70 % se produisent en présence d'un témoin ; un tiers des victimes ont moins de 55 ans ; le taux de survie en France est actuellement de 5 % à 7 %. Certains pays nordiques, mieux formés aux premiers secours, affichent des taux de survie supérieurs à 20 %. En France, si nous parvenions à porter le taux de survie de 7 % à 12 %, voire à 15 %, nous pourrions sauver chaque année 3 000 vies. C'est l'objectif ambitieux fixé par le Président de la République et le Gouvernement d'ici à la fin du quinquennat. Nous ne pouvons qu'y souscrire, À l'heure actuelle, seulement 30 % de la population française est sensibilisée aux gestes qui sauvent, ce qui est bien trop peu, même si l'on note une progression. Chaque année, près d'un million de nos compatriotes s'y initient, principalement par les formations « Prévention et Prévention et secours civiques de niveau 1 » et « Gestes qui sauvent », mises respectivement en place en 2007 et 2017. Et je ne doute pas, monsieur le secrétaire d'État, que le service national universel prendra toute sa part dans la sensibilisation des jeunes. Des modules y seront en effet proposés, en complément des formations dispensées au collège. En outre, l'utilisation des défibrillateurs s'est graduellement répandue. Leur utilisation par le public a été autorisée en 2007, et 180 000 appareils sont installés à ce jour sur le territoire. De plus, la loi du 28 juin 2018 a créé une obligation d'installation d'un défibrillateur automatique visible et d'accès aisé dans certains lieux recevant du public. C'est un sujet qui avait été particulièrement porté par Jean-Pierre Decool, élu à l'Assemblée nationale en 2002, comme moi, et élu sénateur en 2017. Je signale aussi les efforts de nombreuses collectivités pour mettre à disposition des défibrillateurs à proximité des lieux de vie. En dépit de ces progrès, le cadre normatif de la lutte contre les décès par arrêt cardiaque soudain n'est pas encore abouti. La question du régime de responsabilité applicable aux citoyens intervenant pour réanimer les personnes concernées présente des failles et des incertitudes, qui sont de nature à dissuader la prise d'initiative. Des innovations sont à signaler dans ce domaine ; elles s'appuient sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages numériques. Je pense particulièrement à l'application « SAUV life », créée par le SAMU, qui alerte des volontaires quand une personne fait un malaise près de l'endroit où ils se trouvent. S'il est donc souhaitable de faire évoluer la loi, il nous faut tout autant transformer notre culture du secourisme, lequel a trop longtemps été considéré comme un domaine d'expertise et un champ d'action complexe réservé aux bénévoles les plus aguerris et aux professionnels des services d'urgence. La présente proposition de loi a donc pour objectif de porter à l'attention du public la problématique de l'arrêt cardiaque inopiné, et d'encourager les citoyens à se former et à pratiquer les gestes qui sauvent. Bien sûr, ce texte va évoluer, et il est envisageable de penser qu'à l'occasion de la navette parlementaire nos collègues de l'Assemblée nationale n'entendent pas la rigueur juridique dont a fait preuve la commission des lois, et plus particulièrement notre rapporteur, dont je salue le travail. Néanmoins, je suis convaincu qu'il y a des textes sur lesquels nous pouvons et nous devons dépasser les clivages partisans. C'est le cas de cette proposition de loi, issue de la majorité En Marche. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. En conclusion, permettez-moi d'avoir une pensée pour pour l'ensemble de nos services de secours, qui, au quotidien, font un travail remarquable, qu'ils engagent sur le terrain des professionnels ou des bénévoles. Cela inclut, bien sûr, les services départementaux d'incendie et de secours, qui sont, dans nos campagnes, les premiers acteurs dispensant les gestes qui sauvent. Comme ancien président de département, j'ai pu mesurer à quel point nous pouvons compter sur leur engagement et leur courage. À tous nos concitoyens qui sont en première ligne et agissent quotidiennement pour sauver des vies, je dis « merci ! », comme je vous dis « merci de votre attention

: La parole est à M. Jean-Luc Fichet. Il s'agit, par cet amendement, de déterminer qui est le sauveteur occasionnel et bénévole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est un citoyen. Le terme de citoyen permet de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale. La citoyenneté permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société et de participer à la vie politique. Elle donne accès à l'ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs, leur conjonction permettant de participer à la vie civique d'un pays. Dans une société démocratique, la citoyenneté est également l'une des composantes du lien social.

cadre d'application plus général, qui serait relatif à l'ensemble des personnes concourant, par leur comportement, à la sécurité civile, et non plus seulement à celles qui portent assistance à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Au sein de l'armature de ce cadre général, le sauveteur occasionnel et bénévole pourra, en l'espèce, bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public,

et pénale que l'obligation de prévenir les services de secours et de prendre les premières dispositions. Ainsi, la qualité de collaborateur occasionnel ouvrira indistinctement à ses bénéficiaires, quelles que soient les situations auxquelles ils sont confrontés, un certain nombre de protections. Lorsqu'un dommage résultera de leur intervention, leur responsabilité civile ne sera engagée qu'en cas de faute personnelle. Ensuite, nous avons pris le soin d'isoler, dans l'article du code de la sécurité intérieure ainsi amendé, le statut de sauveteur occasionnel, sans lui octroyer pour autant de garanties sectorielles. Enfin, nous avons souhaité préciser que le péril grave et imminent doit être apparent, et non pas forcément établi, afin de ne pas décourager les volontés et de s'aligner, en toute logique, sur l'état actuel de la jurisprudence. L'amendement

non pas seulement au sauveteur occasionnel.

qui tend à rétablir le droit en vigueur, selon lequel les obligations d'appeler les secours et de prendre les premières dispositions sont applicables à toute personne, et non pas seulement au sauveteur occasionnel.